Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Monsieur le président, madame la Première ministre, mes chers collègues, l'évidence est là : l'inflation galope, jusqu'à 7 % d'ici à la fin de l'année, tandis que le pouvoir d'achat des Français recule de 2,9 % sur les premiers trimestres. L'évidence, c'est que les Français les moins aisés souffrent. Bientôt, ce n'est plus de pouvoir d'achat qu'il faudra parler, mais de pouvoir de vivre. L'évidence, c'est que, en 2021, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 174 milliards d'euros de bénéfices, explosant le record, atteint en 2007, de 100 milliards 80 milliards d'euros de dividendes ont été reversés aux actionnaires, ces gens qui profitent du travail des autres, et les salaires des patrons ont augmenté de 23 %. Ce fut l'occasion d'une petite valse du « en même temps » pour Emmanuel Macron, qui dénonçait lors du dernier G7

S'il y a des gens qui tirent des profits de la crise, on souhaiterait que cela puisse bénéficier à tout le monde. » Et vous précisiez que nous n'étions pas dans la situation de nos voisins qui ont instauré une taxe sur les superprofits. « Superprofits », le mot est lâché

une aumône de 20 centimes ou une remise de 250 euros par transport de containers. Nous exigeons une contribution par l'impôt, qui, pour autant qu'il soit juste, est un pilier de la République ! C'est non pas aux conseils d'administration qu'il revient de décider de la participation des entreprises à l'effort national, mais au Parlement, en inscrivant

tout d'abord, nous venons d'apprendre le décès d'un adjudant-chef engagé dans la lutte contre un feu de forêt à Tarascon. Je souhaite lui rendre hommage, adresser toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches

il serait choquant, alors que l'inflation est forte, que certaines entreprises accroissent leurs profits et ne contribuent pas à aider les Français.

préféré mettre les entreprises face à leurs responsabilités et obtenir des résultats concrets. C'est ainsi que TotalEnergies a annoncé une remise de 20 centimes d'euros sur les carburants et que nous avons obtenu de la CMA-CGM une baisse des prix du transport des containers. Ce sont des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des Français. Je crois également qu'un engagement dans la durée est préférable à une taxation ponctuelle. Tel est le sens des mesures que nous vous proposons dans les textes sur le pouvoir d'achat. Nous permettons en particulier aux entreprises d'accompagner leurs salariés face à la hausse des prix du carburant en doublant le plafond de la prime transport. Nous attendons également des entreprises qu'elles soutiennent les revenus de leurs salariés, notamment en se saisissant de la prime de partage de la valeur et des dispositifs d'intéressement et de participation. Enfin, nous demandons à toutes les branches

prenne ses responsabilités, et nous serons prêts à agir s'il le faut dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. La parole

Nous sommes convaincus que notre pays sera capable d'organiser ce grand événement international, qui doit être pour chaque Français et pour chaque Française un moment de fierté. Nous savons que les retombées de ces jeux seront immenses. Les attentes sont donc légitimes et aussi fortes en métropole que dans les outre-mer. À l'issue du conseil olympique et paralympique, le chef de l'État a eu raison d'exiger que tout soit mis en oeuvre pour répondre à cette ambition nous savons tous très grande. Parce que le Gouvernement accorde la même importance aux jeux Olympiques et Paralympiques, nous organiserons deux cérémonies d'ouverture,

Ils attendent également que, contrairement à ce qui s'est passé pour les éditions précédentes, les budgets soient respectés, tant celui du comité d'organisation des jeux que celui de l'établissement public qui assure la construction des sites, en dehors bien entendu des effets de l'inflation, dont personne ici ne pouvait prévoir l'intensité il y a quelques mois encore. Ils espèrent enfin que nous saurons faire de cet événement un levier pour favoriser la pratique sportive au quotidien, dont toutes les études démontrent les effets positifs sur la santé, notamment pour ceux qui en sont aujourd'hui trop éloignés. Madame la Première ministre, comment le comment le Gouvernement entend-il garantir la sécurité des jeux et la qualité des équipements, tout en s'assurant de faire vivre ces jeux pour toutes les Françaises et tous les Français ? La parole Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président Patriat, effectivement, les jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement exceptionnel pour notre pays,

Nous avons réalisé un bilan d'étape et identifié des points de vigilance. Le premier, vous l'avez évoqué, est la sécurité. Sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, les jeux mobiliseront chaque jour entre 7 000 et 11 000 membres des forces de sécurité intérieure. À leurs côtés, interviendront des militaires dont les missions seront précisées en lien avec le ministre des armées, ainsi que des agents de sécurité privés. En lien avec Olivier Dussopt, nous allons intensifier la mobilisation et les formations dans ce secteur, où trop d'emplois demeurent non pourvus. Notre deuxième point d'attention est le budget des jeux.

troisième point est la mobilité. Nous veillerons, avec les collectivités, à garantir le bon déplacement des athlètes et des spectateurs, tout en minimisant leurs conséquences sur le quotidien des Franciliens. Enfin, monsieur le président Patriat, vous avez raison de rappeler que ces jeux doivent être ceux de tous les Français. Ils doivent être porteurs d'un héritage fort pour notre pays

à l'heure de l'hyperconcentration des médias privés et de la concurrence sauvage des grandes plateformes américaines, au lieu de renforcer notre service public de l'audiovisuel, vous avez vous avez décidé de l'affaiblir structurellement et de remettre en cause son indépendance, en supprimant la redevance et en bricolant un financement non pérenne et payé par tous les Français, y compris les plus pauvres : une part fléchée de la TVA que vous retirez à d'autres services et un fléchage qui ne sera plus possible dès 2025. Mes questions sont précises : quels sont les services aux Français qui seront amputés de ces 3,7 milliards d'euros de TVA ? Comment l'audiovisuel public sera-t-il financé à partir de 2025 ?

Nous demandons depuis longtemps une modernisation de la redevance. Pendant cinq ans, vous n'avez rien fait, alors que nos voisins l'ont réformée sans jamais la supprimer. Nous voulons qu'elle soit plus juste et proportionnelle ; vous proposez un financement par l'impôt le plus injuste, à savoir la TVA. Nous voulons qu'elle soit pérenne ; vous proposez un financement dont la fin est formellement programmée en 2025. Si vous étiez ouverts, vous retireriez cette proposition, et nous pourrions mener un travail commun pour la réformer ensemble, dès le budget 2023, à l'automne. En attendant,

ce qui affecterait potentiellement près de 400 000 élèves et familles, et ce dès le mois de septembre prochain. Comme dans beaucoup d'autres métiers difficiles et mal payés, la désaffection ne date pas d'hier. La baisse des vocations a commencé il y a plusieurs années et elle s'est aggravée avec la pandémie. Aux faibles rémunérations, aux horaires décalés et morcelés, s'est ajoutée la fermeture des établissements scolaires pendant la crise du covid. Cela a poussé un grand nombre de personnes à retourner ou à se tourner vers le transport routier de marchandises ou

Au-delà des difficultés propres à chaque métier se posent deux questions : celle de la valorisation de ces personnels, qui nous sont absolument indispensables, et celle du soutien aux élus locaux, qui se démènent pour offrir à nos enfants un accueil approprié. Ces deux questions ne trouveront de réponse que si des mesures d'ampleur sont mises sur la table. Or, en matière de mesures d'ampleur, vous admettrez que c'est bien l'État qui a la main. Certes, les régions s'investissent. Dans le Grand Est, le conseil régional et les rectorats prévoient par exemple d'étaler les horaires de début et de sortie des cours des collèges et des lycées dans six départements, pour qu'un même chauffeur puisse réaliser plusieurs rotations. Mais vous comprendrez bien

Cela passe par des initiatives locales, vous l'avez dit, pour permettre à un même chauffeur de réaliser plusieurs tournées de ramassage scolaire. Cela passe également par la mobilisation du service public de l'emploi, pour recruter, former et sensibiliser sur ce métier, mais aussi pour lui redonner de l'attractivité. Cela passe enfin par des formations.

ma détermination à protéger les Français est totale. Je veux être très clair : toute personne souhaitant être vaccinée contre la variole du singe le sera. Face à cette infection, nous agissons activement. Nous rappelons les gestes de prévention et nous déployons la vaccination, qui est une solution complémentaire à la prévention. Combien y a-t-il de vaccins ? La France a été l'un des premiers pays à ouvrir la vaccination préventive, dès que l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS) a été publié. Je rappelle que celle-ci est gratuite. Plus de 110 centres de vaccination ont été ouverts en seulement quelques jours sur l'ensemble du territoire national.

Nous continuons à monter en puissance. Nous venons par exemple d'ouvrir aux étudiants en santé la possibilité de renforcer les équipes de vaccination pour faciliter l'accès aux rendez-vous. Par ailleurs, un grand centre de vaccination a été ouvert hier dans le XIII arrondissement de Paris, l'Île-de-France étant la région la plus touchée.

toutefois rassurer les Français : 42 000 doses ont été à ce jour déstockées. Les stocks seront libérés au fil de l'eau. De nouvelles commandes de vaccins contre la variole ont été passées tout récemment auprès du seul laboratoire qui produit aujourd'hui ce vaccin de troisième génération, car il faut effectivement poursuivre le renouvellement des stocks. Enfin, même si la variole du singe se diagnostique le plus souvent et très généralement par un examen clinique, il arrive qu'un test biologique soit nécessaire pour compléter le diagnostic. Un arrêté sera publié d'ici à la fin de la semaine, qui permettra une prise en charge de ce test par l'assurance maladie, comme le recommande la HAS. J'ajoute que ma

la secrétaire d'État chargée de l'Europe, en France, chaque village a son église, et chaque église ses vitraux. Ces créations, qui datent souvent de plusieurs siècles, illuminent le patrimoine de tous nos territoires. C'est particulièrement vrai dans l'Aube, où l'on compte la plus grande concentration nationale de vitraux, avec 9 000 mètres carrés de verrières répartis dans 200 édifices. On peut y admirer l'évolution de cet art, du XII siècle à nos jours. Les maîtres verriers sont les dépositaires de ses savoir-faire pluriséculaires. Ils les font vivre par la restauration des vitraux, mais aussi par des créations nouvelles, qui excèdent largement le cadre religieux. Or, pour continuer à faire vivre ces savoir-faire de restauration et de création, les vitraillistes ont depuis toujours recours au plomb. Cette substance, dont la toxicité est avérée, est intégrée à leur pratique. Ils s'en protègent les

c'est bien simple : si le plomb est interdit, les vitraillistes ne pourront plus exercer leur activité. Pour prendre un exemple concret qui parle à chacun d'entre nous, sans plomb, il serait impossible de restaurer à l'identique les vitraux de Notre-Dame de Paris. J'ai déposé une proposition de résolution européenne pour défendre cette exemption, de droit et sans frais, pour tous les vitraillistes. Le Sénat l'a adoptée. Je tiens d'ailleurs à remercier les deux rapporteurs qui ont planché sur ce texte, mes collègues Catherine Morin-Desailly et Louis-Jean de Nicolaÿ, qui ont montré que d'autres métiers d'art, tels les facteurs d'orgues, étaient également menacés par cette interdiction. Madame la secrétaire d'État, ma question est simple : défendrez-vous à l'échelon européen une exemption à titre gracieux pour ces métiers d'art ? La chambre des territoires vous le demande. Il y va de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine exceptionnel. La parole Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Paoli-Gagin, votre question me donne l'occasion de vous remercier du travail réalisé depuis plusieurs semaines sur cet enjeu important

soumises à autorisation. Le Gouvernement a entendu la voix du Sénat sur ce sujet. Je puis vous assurer de notre pleine mobilisation auprès de la Commission européenne pour garantir que toute évolution de la réglementation en la matière permettra de préserver l'ensemble du secteur du vitrail, des monuments historiques et du patrimoine culturel. La parole est à M. Mathieu Darnaud, pour le groupe Les Républicains.

à la revalorisation de 3,5 % du point d'indice dans la fonction publique ou encore à l'inflation galopante. La réponse du Gouvernement est quelque peu déconcertante. Le 7 juillet dernier, lors d'une réunion de la commission des finances, votre éminent collègue Bruno Le Maire

d'apaiser les inquiétudes légitimes des élus locaux, qui, comme les ménages, s'interrogent, dans un contexte d'inflation forte, et se trouvent confrontés à une équation simple : les dépenses augmentent, nous sommes collectivement hostiles à l'augmentation des impôts et nous considérons dans le même temps que la dépense publique est un sujet sérieux.

Monsieur le ministre, le flou se nourrit aussi de ce que l'on ne dit pas. En l'occurrence, vous avez indiqué ce que vous ne ferez pas, mais vous n'avez pas dit ce que vous comptiez faire. Vous n'avez surtout avancé aucun chiffre,

ce document laisse plutôt songeur : entre 2013 et 2020, ce sont 19 000 lits qui ont été supprimés à l'hôpital public. Plus problématique encore, ces fermetures se sont accélérées en 2020, en pleine crise du covid : au total, 5 700 lits ont été fermés cette année-là, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 2019, alors qu'elle était jusque-là, en moyenne, de 0,9 % par an. Rien ne justifiait une accélération aussi insensée, sinon un virage net vers l'ambulatoire et la perpétuation de mesures budgétaires prises bien avant la crise. L'hôpital s'est recentré sur sa vocation d'urgence. La pandémie a entraîné une hausse significative des capacités en soins critiques. Pour le reste, on compte sur la médecine de ville, sans s'assurer que la prise en charge soit possible ... C'est nier que l'activité hospitalière déborde largement le cadre de l'urgence. En parallèle, malheureusement, les capacités ambulatoires ne sont pas adaptées à due proportion. Monsieur le ministre, la fermeture de lits ouvre un cercle vicieux de pénurie de personnel. Moins de lits, c'est moins de personnel, ce qui entraîne en retour la fermeture de nouveaux lits. Dans ces conditions, le virage vers l'ambulatoire ne peut s'analyser que comme une mesure financière, et non comme une politique sanitaire. Monsieur le ministre, à rebours des différents plans encore en cours, cesserez-vous enfin les fermetures définitives de lits à l'hôpital ? Mettrez-vous fin

De plus, durant la crise du covid, nous avons dû procéder à des réorganisations : pour éviter la contagion, des chambres doubles ont dû être transformées en chambres simples, réduisant de fait le nombre de lits. De nombreux lits ont été ouverts en soins critiques.

Tel sera l'objet de la concertation des parties prenantes, qui doit nous permettre de trouver des solutions pragmatiques, applicables sur le terrain, en fonction des besoins identifiés de chaque territoire. Je m'appuierai également sur le travail des parlementaires. La parole est à Mme

La presse quotidienne régionale nous informe de ces attaques. Pour les derniers jours, il faut citer Angers, Amiens, Montpellier, Loriol-sur-Drôme, Metz et tant d'autres communes qui ont connu ces drames. Ces attaques au couteau sont parfois le fait d'étrangers déjà connus défavorablement des services de police, ce qui nous plonge dans l'incompréhension.

Vous évoquez des étrangers en situation régulière ou irrégulière qu'on laisserait libres de commettre des actes délictuels ou criminels. Je me suis exprimé très clairement à ce sujet et je rappelle que, depuis deux ans, nous avons expulsé 3 000 étrangers délinquants.

formulées, alors qu'elles ont été rejetées avec mépris sous les quinquennats Hollande et Macron. Les peines planchers pour ceux qui attaquent nos forces de l'ordre ? Rejetées ! Les places de prison supplémentaires ? Nous attendons encore. L'expulsion des étrangers qui représentent une menace

Quel manque d'anticipation, surtout ! Les personnes recrutées lors de ces séances de exerceront demain devant vos enfants et petits-enfants, mes chers collègues, sans formation, plongés dans le bain bouillonnant des classes, au hasard, selon une statistique inconnue et aléatoire. Les enfants de la République méritent mieux que cela. Enseigner est non seulement une vocation, mais surtout un métier, qui ne s'improvise pas. Enseigner nécessite tout à la fois des qualités personnelles indispensables et une formation solide. Constat amer, le métier de professeur n'est plus attractif,

Être civilisé, n'est-ce pas assurer l'accès au savoir et à la connaissance et permettre à tous les enfants de France, comme cela a été le cas pour vous, monsieur le ministre, de devenir ce qu'ils doivent être ? Il y a parmi les étudiants pauvres des vocations qui ne se réalisent pas.

de certains concours de recrutement des enseignants, phénomène relevé récemment dans un rapport très informé du sénateur Gérard Longuet. Nous sommes cette année confrontés à une situation un peu particulière, du fait, tout d'abord, de la réforme engagée pour

Au regard de cette situation, le ministère a mis en place une série de mesures pour assurer les meilleures conditions de rentrée possible, dont des recrutements sur liste complémentaire, des concours supplémentaires et des recrutements d'enseignants contractuels, qui ne se font pas du tout en quelques instants ni selon les termes que vous avez décrits, madame la sénatrice. L'objectif reste que tous les élèves soient accueillis et qu'un professeur soit présent devant chaque classe.

pour prévenir et résoudre les dernières difficultés. Enfin, conformément aux engagements du Président de la République et de la Première ministre, la revalorisation à venir dans le cadre du pacte avec les enseignants fera l'objet d'une concertation pour renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement, mieux reconnaître l'engagement de chacune et chacun des professeurs et pour repenser finement les dynamiques et les évolutions de carrière.

malheureusement pour moi, c'est le treizième depuis que je suis élu parisien. Vous avez défini un ordre de mission précis, très complet, qui est en même temps un bilan des insuffisances de l'institution et des déficiences de la sécurité à Paris.

On ne compte plus les vagues caniculaires qui s'abattent sur le territoire, toujours plus précoces, toujours plus fréquentes et toujours plus intenses. Le 25 juillet dernier, nous apprenions que la quasi-totalité des départements de France étaient concernés par des restrictions d'utilisation de l'eau : pas moins clairs, la sécheresse est là. De plus, avec la hausse massive des températures, le phénomène d'évapotranspiration des plantes augmente et le bilan hydrique des sols devient alarmant. L'eau est un enjeu majeur pour le monde agricole. Sans mobilisation des pouvoirs publics, c'est notre agriculture tout entière qui sera menacée. Or, face à ce fléau, nos agriculteurs se sentent abandonnés. Leur situation est déjà très difficile, et il est de notre devoir de continuer à les aider. Il nous faut absolument développer nos efforts pour capter l'eau. En effet, monsieur le ministre, le problème n'est pas tant l'eau que sa captation et sa gestion tout au long de l'année. L'agence de l'eau Adour-Garonne prévoit même que le volume de pluie annuel sera plus important d'ici à 2050 qu'il Des solutions existent, comme les retenues collinaires ou les barrages, mais elles sont difficiles à mettre en oeuvre. Les normes bloquent et découragent toute initiative en ce sens. Vous me répondrez sans doute que le problème vient de l'Europe. Mais alors, pourquoi l'Espagne, qui a deux fois moins de ressources en eau que la France, parvient-elle à en capter presque dix fois plus ? Pour y arriver, il faut du volontarisme et du courage politique. Or l'État en a souvent manqué durant ces dernières années. L'abandon du barrage de Sivens en est un exemple caractéristique. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer concrètement quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour aider le monde agricole à faire face aux épisodes de sécheresse ? La parole

En effet, les procédures d'expulsion, lorsqu'elles sont engagées, tardent à être mises en oeuvre et se révèlent inefficaces. Tout à fait ! De tels retards ont des conséquences environnementales, économiques et sanitaires extrêmement dommageables

Ma question est donc la suivante : face au désarroi de nos administrés, de nos élus et de nos forces de l'ordre, et avant qu'un drame ne se produise, qu'envisagez-vous de faire, monsieur le ministre ? Il y a urgence.

Monsieur le ministre, nos communes ne doivent plus souffrir à cause d'une minorité qui ne respecte pas les lois de la République. Néanmoins, face au contexte si tendu que je décrivais, et pour faire suite aux propos de Mme la Première ministre Élisabeth Borne, qualifiant le Sénat de « chambre d'apaisement et d'équilibre », je vous invite à soutenir la proposition de loi de mes collègues Patrick Chaize, Sylviane Noël et Alain Chatillon, votée ici même et visant à consolider les outils juridiques permettant aux maires de mettre fin aux occupations illégales des gens du voyage. La

En France, rien ! Nous sommes assis sur le banc des mauvais élèves. Malgré un afflux de 1,4 million de billets longue distance vendus seulement pour les mois de juillet et d'août, malgré une inflation qui rend la situation des Français

Pourtant, la planète a besoin de plus de trains ; les citoyens ont besoin de prix plus bas ; la SNCF a besoin de plus d'argent. Et, monsieur le ministre, vous rejetez la faute sur les Français. Vous les invitez à réserver leur billet en avance, grâce à des cartes de réduction en choisissant les horaires moins coûteux. Insinuer ainsi que les citoyens achètent volontairement les billets les plus chers témoigne de votre déconnexion et de votre incompréhension des difficultés des Français

concentrer l'effort budgétaire, politique et territorial, dans les prochains mois, pour la réplique. C'est un fait, monsieur le ministre : tout ce que vous avez pu mettre en oeuvre n'a visiblement pas eu de conséquences sur le prix des billets, donc sur le pouvoir d'achat des Français.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement a mis en place, depuis novembre 2021, un bouclier tarifaire afin de limiter la hausse des prix de l'électricité et du gaz à 4 %. En effet, les coûts de l'énergie explosent, et les Français doivent pouvoir payer leurs factures. Cette mesure est à saluer, puisque, sans son adoption, les prix auraient augmenté de 45 %.

Leur situation est pourtant identique à celle de l'ensemble des particuliers, puisqu'ils résident dans un lieu d'habitation, selon un contrat de prestations à durée indéterminée, sur lequel figure aussi la fourniture d'énergie.

de ma commune de Gerstheim, des calculs prévisionnels montrent que l'augmentation pourra atteindre jusqu'à 469 % pour les heures pleines hiver, sans compter les taxes.

comme une parfaite concrétisation du discours de la méthode de Mme la Première ministre ? Monsieur le ministre, profiterez-vous du silence législatif de l'été pour échanger sur un projet de loi de finances initiale pour 2023 sécurisé parce qu'inscrit dans une trajectoire pluriannuelle,

nous avons une chef, et elle a défini un cap, ici, à la tribune du Sénat à l'occasion de sa déclaration de politique générale. Fayot ! Ce cap, c'est celui de la coconstruction. Le 19 juillet dernier, lorsque j'ai reçu les associations d'élus,

des balises que j'ai eu l'occasion de rappeler et que le sénateur Mathieu Darnaud a parfaitement retenues, concernant notamment l'absence de baisse des dotations des collectivités territoriales- l'absence totale de ponction,

Monsieur le ministre, quitte à m'attirer les foudres de mes collègues, je salue votre chef, ainsi que sa méthode ! Je salue aussi le mien, qui nous invite

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Mes chers chers collègues, si les pouvoirs publics font des efforts, depuis la grande canicule de 2003, afin de lancer des campagnes de prévention pendant les pics de chaleur, le système pénitentiaire doit, seul, faire face à à la crise, et les détenus se débrouiller avec le peu de moyens à leur disposition, alors même que la surpopulation carcérale atteint des sommets.

Au dernier étage, dans la coursive à ciel ouvert, la température était de 45 degrés. Des détenus répandaient de l'eau par terre et marchaient pieds nus pour se rafraîchir. Ils parlaient de leur souffrance ; ils demandaient un peu d'humanité, plus de douches et moins de surpopulation pour commencer. Monsieur le ministre, que compte faire l'État pour rénover nos prisons et les adapter au réchauffement climatique ? L'enfer, ce n'est pas les autres, comme Sartre l'écrivait. L'enfer, c'est la prison en temps de canicule. La

en place la semaine dernière ; enfin, permettre davantage de douches que ce que prévoit la réglementation. La prison, on le sait, est faite pour punir

prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 27 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Jean Castex à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. au Gouvernement. Les prochaines questions d'actualité au Gouvernement auront lieu le mercredi 5 octobre 2022,